de l'article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 13 juillet 2017, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière de transports sur le projet de nomination de Mme Catherine Guillouard aux fonctions de président-directeur général de la RATP. Cette demande d'avis a été transmise à la commission de l'aménagement du territoire. Acte est donné de cette communication. J'informe le Sénat que le groupe Les Républicains a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour remplacer, en qualité de secrétaire du Sénat, M. Christian Cambon. La candidature de M. Jean-Paul Émorine a été publiée et la désignation aura lieu conformément à l'article 3 du règlement. Très bon candidat ! La parole est à M. Bernard Delcros.

à la demande notamment de M. le président Guillaume. Le président du Sénat a envisagé, avec le Gouvernement, la possibilité de siéger, le cas échéant, lundi à partir de

la discussion se déroule dans les meilleures conditions possible, avec des prises de parole concises. Très bien ! Tout dépendra éventuellement du vote sur les amendements de suppression de l'article 9.

aujourd'hui, grâce au règlement du Sénat et à l'action de la commission des finances, en particulier de sa présidente, la répartition de la réserve parlementaire est transparente et très claire. Je suis sénatrice du Pas-de-Calais, soit un département qui compte plus de 700 communes rurales. Je puis vous dire que l'ensemble des sénateurs du Pas-de-Calais, tous engagements partisans confondus, répartit la réserve parlementaire de façon égalitaire, en fonction des projets proposés

sauf amendement de suppression pur et simple. Ce n'est évidemment pas le meilleur moyen de promouvoir une relation constructive entre le Parlement et le Gouvernement

au-delà des abus auxquels il était indispensable de remédier, la réserve remplissait une fonction extrêmement utile, non seulement en France, en faveur essentiellement des toutes

Il appartient à l'État et aux exécutifs locaux de conduire des politiques publiques par le biais d'un budget qui sera voté par le Parlement ou par l'assemblée délibérante,

attribué aux collectivités locales au titre de la réserve parlementaire, soit 86 millions d'euros, soit réorienté vers les territoires.

des lois. L'inscription dans la loi organique relative aux lois de finances d'un mécanisme clairement défini constitue, à n'en pas douter, un progrès par rapport à la situation actuelle de la réserve parlementaire, qui est un non-dit budgétaire et juridique.

Toutefois, j'ai le sentiment que nous avons encore besoin d'un peu de temps pour avancer dans l'écriture de ce texte et que le travail que le Gouvernement sera amené à conduire avec l'Assemblée nationale nous permettra, sur la basse de la piste que vous avez ouverte, d'aller

Il s'agit de maintenir la dotation et de la centrer sur l'investissement des communes et sur les associations, en limitant le volume des fonds

En effet, ce texte prévoit un dispositif de soutien à l'investissement des communes et des groupements de communes. De fait, ne sont pas inclus les organismes qui, hors hexagone, sollicitent les sénateurs représentant les Français établis hors de France

En France, le maillage administratif permet d'identifier les besoins et de trouver différents moyens d'y répondre. À l'étranger, malheureusement, ne se trouvent que des consulats qui représentent l'administration française et qui ne disposent pas de crédits pour répondre à ces demandes, à la seule exception de crédits d'aide à la personne prenant la forme de bourses scolaires ou d'aides sociales. nous, il convient de maintenir la possibilité, pour les parlementaires, d'aider ces organismes de toute nature qui oeuvrent en faveur du rayonnement de notre pays à l'étranger. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, je vous propose d'adopter cet amendement.

Nous refusons la suppression de la réserve parlementaire sans que soit reconstituée une forme de dotation de l'État qui pourrait financer les projets soumis à l'État par les parlementaires.

que de demander purement et simplement sa suppression. D'accord ! Nous serons plus forts pour dire au Gouvernement que nous voulons maintenir un système de financement pour les communes rurales, avec fléchage

pour cinq raisons. Vous en souhaitiez une, monsieur Delcros, je vous en donne cinq ! Premièrement, la réserve ministérielle sert à subventionner des dossiers d'investissement des collectivités locales qui sont liés à des dépenses exceptionnelles. Elle est donc très

Quatrièmement, à titre principal, ces crédits sont inscrits dans le projet de loi de finances au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », dans le programme 122 « Concours spécifiques et administration ».

acceptable que les parlementaires fassent l'objet d'une défiance si grande qu'on inventerait pour eux une procédure particulière, alors qu'ils sont élus et ont des comptes à rendre à la Nation, tandis que les

monsieur le rapporteur

encadrement de la réserve parlementaire, suppression des emplois familiaux, amélioration du statut des collaborateurs parlementaires, réflexion sur l'accès au financement des candidats et partis politiques. Surtout grâce au travail du Sénat ! Reste que ne sont pas abordés des points essentiels, qui expliquent la perte de confiance de nos concitoyens dans le système politique. La lutte

qui visaient des points ayant pourtant un lien direct, comme l'exige l'article 45 de la Constitution, avec ces projets de loi ordinaire et organique. Aucun ! Restaurer la confiance, c'est aussi permettre le débat. Moraliser les rapports entre médias, politique et argent n'a-t-il aucun lien avec le rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans la vie publique ? Améliorer la représentativité des parlementaires en instaurant la proportionnelle, cela n'a-t-il aucun lien avec le rétablissement de la confiance dans l'action publique ? Cesser le ballet indécent et permanent des sondages organisés par des entreprises et officines en lieu et nom de la politique et de l'argent, cela n'a-t-il aucun lien avec le rétablissement de la confiance ? Et encore, madame la garde des sceaux, nous ne nous sommes pas attaqués à la moralisation de l'économie et à l'absence d'intervention de la puissance publique pour rappeler à l'ordre le monde de l'argent, qui piétine l'intérêt général en permanence ! Ces projets de loi ont un double objectif : tenter de répondre au ras le bol de nos concitoyens tout en ne touchant pas à cette question de fond, l'intrusion massive de l'argent dans la politique. C'est pourquoi, malgré l'adoption de trois de nos amendements- suppression du verrou de Bercy, inscription, contre l'avis du Gouvernement, de l'abus de bien social comme motif d'inéligibilité, accès au concours interne de la fonction publique

Le débat y est riche. Nos concitoyens y sont très attentifs. Il est impératif qu'ils comprennent mieux notre travail et qu'ils puissent y contribuer. C'est essentiel dans l'oeuvre de reconnexion démocratique

compromis qui a été trouvé par la commission des lois et son président sur la réserve parlementaire. Il fallait vraiment trouver une solution,

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

a présenté la candidature de M. Jean-Paul Émorine pour remplacer, en qualité de secrétaire du Sénat, M. Christian Cambon. Très bonne candidature ! Le délai prévu par l'article 3 du règlement est expiré. La présidence n'a reçu aucune opposition.

le Sénat accueillera la journée de lancement de la Conférence nationale des territoires. À cette occasion, le président du Sénat recevra le Président de la République et le Premier ministre. à quatorze heures trente en salle Clemenceau par un discours du président du Sénat, qui sera suivi d'une intervention du Président de la République. Tous les sénateurs sont conviés à cet échange, qui se prolongera par des ateliers thématiques.

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (procédure accélérée)